La nomination des officiers supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires a été déconcentrée au niveau départemental, ce qui est une bonne chose. Par voie de conséquence, la Commission nationale, qui était chargée jusqu'alors d'émettre un avis sur les propositions des SDIS, a été supprimée. les effets de cette suppression et d'évaluer l'impact de cette déconcentration, cet amendement vise à prévoir la présentation par le Gouvernement d'un rapport annuel au Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires en vue d'opérer le suivi, l'évaluation et l'impulsion nécessaire, pour assurer l'accès effectif des sapeurs-pompiers volontaires à l'encadrement opérationnel et fonctionnel des SDIS. L'amendement

: La parole est à Mme Émilienne Poumirol. Il convient de prévoir la présentation par le ministère de l'intérieur d'un rapport annuel au Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, afin d'opérer le suivi, l'évaluation et l'impulsion nécessaire à l'accès effectif des sapeurs-pompiers volontaires à l'encadrement opérationnel et fonctionnel des SDIS. telle disposition est motivée par la concentration à l'échelon départemental de la nomination des officiers supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires, qui entraîne de fait la suppression de la Commission nationale chargée d'émettre un avis sur les propositions des SDIS. En vous soumettant cet amendement, mes chers collègues, nous nous inscrivons dans la logique du plan d'action de 2019-2021 en faveur du volontariat, que le Gouvernement a présenté le 29 septembre 2018. Ce dernier vise trois objectifs essentiels attirer et susciter des vocations, en représentant mieux notre société, en donnant toute leur place aux femmes et en intégrant les jeunes de tous les horizons ; fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires et les mettre au coeur du dispositif, en prenant en compte leurs compétences individuelles,

Ces trois amendements sont contraires à la position de la commission, qui y est donc défavorable. Ils visent à instaurer un rapport annuel remis par le ministère de l'intérieur au Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et consacré au suivi et à l'évaluation de l'accès des sapeurs-pompiers volontaires à l'encadrement opérationnel et fonctionnel des SDIS. Il est certes important de favoriser cet accès. Toutefois, nous ne sommes pas convaincus de l'intérêt ni du caractère opérationnel des rapports annuels de suivi.

La présente proposition de loi transfère la mission d'organisation des concours et examens professionnels des catégories A et B des sapeurs-pompiers professionnels aux centres de gestion, le CNFPT se chargeant, Le transfert aux centres de gestion de la compétence d'organisation des concours et examens professionnels de catégories A et B s'accompagne du versement d'une compensation financière. Cependant, cette dernière ne peut être versée à l'un des centres coordonnateurs désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ; elle doit être versée aux centres de de gestion coordonnateurs dans le ressort desquels les centres de gestion organisent ces concours et examens. Le présent amendement a pour objet de respecter la compétence de chaque CDG en évitant d'ériger l'un des centres coordonnateurs en coordonnateur et gestionnaire d'un ensemble d'établissements publics de même nature, qui méconnaîtrait le principe constitutionnel d'égalité entre établissements publics. Il tend également à reproduire le mécanisme de compensation financière existant

en raison du transfert aux centres de gestion des concours et examens professionnels des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégories A et B. Il convient en effet de respecter la compétence de chaque centre de gestion, ainsi que le principe d'égalité entre des établissements publics similaires, en évitant d'ériger l'un de ces centres coordonnateurs en centre gestionnaire, ce qui reviendrait à attribuer une nouvelle mission à ce centre particulier. En conséquence, l'amendement tend également à remplacer le mécanisme de convention initialement prévu entre le centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion organisateurs par un conventionnement entre l'ensemble des centres de gestion coordonnateurs et les centres de gestion organisateurs de leur ressort. Quel est l'avis du Gouvernement ? Le

la formation des officiers sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et des personnels dédiés doit rester globalement sous la responsabilité du CNFPT, en tant que collecteur des cotisations versées par les SDIS. Le CNFPT est reconnu pour son expertise et forme déjà tous les non-officiers, les sapeurs, les caporaux et les sous-officiers. Il y doit y avoir une unité dans la formation des sapeurs-pompiers, sous l'autorité du CNFPT. Dans ces conditions, il n'est pas utile de réaliser un rapport pour envisager de transférer l'entière responsabilité de la formation des officiers et des cotisations à l'Ensosp. Nous demandons donc la suppression de

L'Ensosp fait aujourd'hui face à des défis structurels : elle ne dispose pas de schéma de financement pérenne ; la répartition des compétences avec le CNFPT mériterait d'être clarifiée ; elle est laissée en dehors de la réforme de la formation de la haute fonction publique ; enfin, sa gouvernance est trop déséquilibrée. La commission a acté la nécessité d'explorer des pistes de réforme pour répondre à ces défis. J'émets donc un avis défavorable

: La parole est à Mme Guylène Pantel. Comme cela a pu être souligné lors de la discussion générale, il est absolument nécessaire, dans les années à venir, de solliciter davantage notre jeunesse, afin de faire naître des vocations pour les fonctions de sapeurs-pompiers. Aussi cet amendement vise-t-il à ajouter une évaluation des dispositifs de formation des jeunes sapeurs-pompiers, qui préfigurent assez souvent un engagement plus définitif dans le corps des sapeurs-pompiers. Les auteurs de l'amendement rappellent par ailleurs que des dispositifs de section d'études de jeunes sapeurs-pompiers au sein de structures scolaires existent, grâce à l'engagement de formateurs de l'école. Ils méritent d'être soutenus et valorisés, en partenariat avec l'éducation nationale. de la commission ? Le rapport évoqué à l'article 19 concerne uniquement la formation des officiers de sapeurs-pompiers et la réforme de l'Ensosp. La formation des jeunes sapeurs-pompiers est bien entendu un sujet majeur, qui doit être étudié avec soin, mais elle ne trouve pas sa place dans ce rapport. Je vous demande donc, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre

Cet enseignement serait par ailleurs l'occasion de mener une politique de prévention associant directement les sapeurs-pompiers volontaires aux enjeux de prévention des risques climatiques que pourraient devoir affronter les plus jeunes dans les prochaines années. Quel est l'avis de la commission ? Le présent ? Le présent amendement tend à préciser, au sein du code de l'éducation, que les élèves bénéficient d'une sensibilisation à l'engagement de sapeur-pompier volontaire durant leur scolarité. Nous sommes très sensibles à cette démarche et à la promotion du volontariat en règle générale. Toutefois, la récente loi dite « Citoyen sauveteur » a rendu obligatoire une sensibilisation « aux missions des services de secours ». Nous pensons qu'elle couvre déjà la sensibilisation au volontariat en tant que composante incontournable des services de secours. La commission demande donc le retrait de cet amendement

: La parole est à M. Jérôme Durain. L'article 21 de la proposition de loi crée un nouveau statut de pupille de la République pour les orphelins des personnes dont l'acte de décès porte la mention Mort pour le service de la République », militaires ou agents publics appartenant à des corps ou entités habituellement exposés à des situations de danger, tels les agents de police, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, les agents des douanes ou de l'administration pénitentiaire, ainsi que les sauveteurs en mer. Cet article important vient concrétiser un engagement du Président de la République. Il permettra à l'État d'exprimer sa gratitude et sa reconnaissance de manière officielle envers ceux qui meurent en service. Il permettra à leurs enfants d'être soutenus et accompagnés en tant que pupilles de la République. Le présent amendement vise à parachever la création de ce nouveau statut, afin de venir en complément des dispositifs qui existent déjà. Nous pensons qu'il est utile de conforter les missions de protection et de soutien matériel et moral apportés aux enfants des sapeurs-pompiers et des personnels de la sécurité civile accomplies par l'OEuvre des pupilles orphelins et Fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France, l'ODP, comme le fait l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les militaires, dans le cadre du statut de pupille. L'ODP

Cette évolution nous a semblé de nature à simplifier la gestion de ce nouveau pupillat, qui serait centré sur les aides apportées par l'État en matières éducative, sociale et fiscale. C'est pourquoi il nous semble pertinent de conserver la création du pupillat de la République. La commission est donc défavorable

d'entraide des sapeurs-pompiers de France l'accompagnement des enfants des sapeurs-pompiers et des personnels de la sécurité civile pupilles de la République. Si nous comprenons l'objectif visé, l'attribution de l'accompagnement des pupilles de la République à tel ou tel organisme relèvera d'une convention entre cet organisme et l'État.

dans la mesure où l'orphelin y est éligible dès lors que son parent a notamment été tué ou est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait d'un événement de guerre ou d'une OPEX, c'est-à-dire dans des circonstances le rendant le rendant éligible à la mention « Mort pour la France ». Peuvent également être pupilles de la Nation les orphelins d'agents publics tués du fait de l'acte volontaire d'un tiers

que les enfants de moins de 22 ans des personnes reconnues mortes « pour le service de la République » du fait notamment de l'accomplissement de leurs fonctions dans des conditions impliquant un danger ou un risque particulier non lié à l'acte volontaire d'un tiers puissent aussi bénéficier de la qualité de « pupille de la République Si les deux statuts de pupilles sont formellement distincts juridiquement, les droits associés à la qualité de pupille de la République sont, par équité pour les orphelins endeuillés par le décès tragique de l'un de leurs parents, très similaires sont octroyés aux pupilles de la Nation, en particulier s'agissant de la matérialité de l'accompagnement qui leur est dispensé et des aides financières qui leur sont légitimement accordées. En outre, le pupillat de la République ne prévoit pas, comme le pupillat de la Nation, une procédure d'adoption devant le juge. Il en résulte, certes, une moindre charge symbolique, mais aussi une plus grande facilité et un délai potentiellement raccourci pour la mise en place de l'accompagnement, cela a été relevé dans tous les travaux préparatoires. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut se voir confier par convention, pour le compte de l'État, l'accompagnement des pupilles de la République. Cette disposition ouvre une possibilité qu'il était indispensable de prévoir explicitement pour que cet opérateur de l'État, avec des missions bien délimitées, puisse se voir confier, pour le compte et par financement d'un ministère autre que celui des armées, le suivi

En effet, le fait d'être pupille de la Nation implique une adoption par la Nation. Si nous comprenons bien la charge symbolique, affective et psychologique que cela peut représenter, nous souhaitions simplement- je pense que nos collègues sont dans le même état d'esprit

de la République pour les enfants des personnes auxquelles cette mention aura été attribuée. Les alinéas 20 à 22, introduits lors de l'examen en commission au Sénat, visent à préciser, au sein de l'article L. 411-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,

de la commission ? Nos collègues du groupe RDPI souhaitent, par leur amendement, supprimer une coordination que nous avons introduite en commission, estimant qu'elle est superflue, car le non-cumul des régimes est déjà prévu par ailleurs. Le principe même des coordinations est cependant de faire en sorte que l'ensemble des dispositions de notre législation soient harmonisées entre elles. Puisque nous sommes d'accord sur le fond du dispositif, je ne vois aucune

des militaires tués en service ou en raison de leur qualité de militaire et, d'autre part, des autres agents publics tués en raison de leurs fonctions ou de leur qualité. L'alinéa 23 de l'article 21, que cet amendement tend à supprimer, ajoute une condition à cette attribution,

La mention « Mort pour le service de la Nation » serait réservée aux personnes tuées parce qu'elles représentaient, dans leur fonction, la République, tandis que la mention « Mort pour le service de la République » acterait la reconnaissance de la France pour l'engagement exceptionnel d'une personne ayant conduit à son décès. Cet effort de distinction me paraît louable. C'est la raison pour laquelle je vous invite, mon cher collègue, à retirer votre amendement.

prime sur le droit français. Ce premier constat nous conduit, comme d'autres collègues ici, à demander la suppression de cet article, pour souligner son absence de portée. La directive européenne sur le temps de travail de 2003 puis la jurisprudence de 2018 appliquent en effet aux pompiers volontaires des règles sur l'aménagement du temps de travail, comme le plafonnement à quarante-huit heures par semaine de l'activité cumulée entre travail et volontariat, le repos de sécurité quotidien et le paiement des cotisations salariales. Nous partageons évidemment l'inquiétude générale face à l'application de ces règles en France, où le statut de pompier volontaire

la discussion générale ainsi que par Cécile Cukierman à l'instant. Je comprends la volonté du Gouvernement de sauvegarder le modèle de volontariat qui est au coeur de l'organisation des pompiers. De nombreuses questions ont été posées, dans cet hémicycle, depuis le début de

l'application de cette jurisprudence au système français de sécurité civile, qui compte, je le rappelle, 80 % de sapeurs-pompiers volontaires, aurait des conséquences insurmontables

relance du volontariat ; et ce rapport était sans appel : « Nous demandons au Président de la République et au Gouvernement d'exprimer une position politique déterminée auprès du Conseil de l'Union et de la Commission européenne pour exempter

il a été largement admis que la mesure proposée à cet article emportait essentiellement un soutien clair au volontariat ; il s'est agi de réaffirmer, par une mesure adoptée à l'unanimité, que l'activité de sapeur-pompier volontaire ne pouvait être assimilée à celle de travailleur. Pour autant, bien sûr, le Gouvernement partage le point de vue des rapporteurs sur le caractère peu opérant de la mesure prévue à cet article. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous nous en remettons à la sagesse

la position de la France sur l'absence d'applicabilité de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, dite DETT. Ainsi l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n'implique-t-il nullement que tout sapeur-pompier volontaire doive automatiquement être considéré comme un travailleur au sens de la DETT- c'est très clair. Néanmoins, ces échanges ne permettent d'offrir des garanties raisonnables pour faire durer notre modèle de volontariat que pour autant que l'on traite les situations locales, minoritaires probablement, qui pourraient le fragiliser devant les juridictions. Il nous semble en effet utile de préciser que ces échanges ne lient en rien la Commission ou une juridiction nationale, alors que des contentieux en sont déjà au niveau de l'appel que certains renvois préjudiciels pouvant avoir un impact sur les activités de sapeur-pompier sont en cours et qu'il nous faut encore agir pour traiter au mieux ces fragilités. Nos services ont lancé une large concertation en ce sens, visant tout d'abord à disposer d'un point précis de situation sur l'organisation du recours au volontariat dans les services d'incendie et de secours, ainsi que sur les propositions concrètes que ceux-ci peuvent faire pour traiter les fragilités qu'ils auraient identifiées. Cet état des lieux, qui est en cours de consolidation, sera suivi par la mise en place de groupes de travail constitués, comme le ministre de l'intérieur s'y est engagé, pour partager les constats et identifier les nouvelles actions correctrices à entreprendre ensemble. À l'issue de ces travaux viendra le troisième temps, celui des ajustements. Ceux-ci n'auront pas vocation à imposer des contraintes inadaptées aux territoires, mais au contraire à poser des bornes acceptables et nécessaires au respect des exigences de l'Union européenne. Vous l'aurez compris, ces mesures doivent être de nature à nous prémunir contre les fragilités évoquées face à de possibles contentieux. Plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, ont évoqué l'occasion que représente la présidence française de l'Union européenne. Je souhaite y revenir brièvement pour dire que la France prendra une initiative pour la valorisation de l'engagement citoyen ; ce travail complémentaire permettra d'asseoir davantage notre modèle de sécurité civile. Comme vous pouvez le constater, le Gouvernement est pleinement engagé, en liaison étroite avec les services d'incendie et de secours et avec l'ensemble des acteurs et partenaires concernés, dans la consolidation de notre modèle de volontariat. Je sais pouvoir compter sur vos analyses et, bien entendu, sur vos propositions. La parole

Si je comprends bien les arguments juridiques et l'objectif louable de la commission, les conséquences de la décision européenne qualifiant les sapeurs-pompiers volontaires de travailleurs seront lourdes pour eux et pour notre système de secours. L'article L'article 22 A a une portée limitée par rapport à la directive européenne. Si le temps d'intervention des sapeurs-pompiers volontaires était comptabilisé dans le temps de travail, cela équivaudrait à supprimer

l'engagement de sapeur-pompier volontaire est un engagement citoyen, librement décidé et consenti, visant à favoriser, à promouvoir et à garantir des activités d'intérêt général ou permettant de satisfaire un besoin social ou sociétal, et plus particulièrement la nécessité de faire face aux risques et aux enjeux de protection publique et de protection civile. Compte tenu des éléments exposés par nos rapporteurs et pour manifester notre soutien à leur proposition, nous retirons cet amendement.

Doineau. La présente proposition de loi se donne pour objectif de consolider notre modèle de sécurité civile, qui repose à plus de 80 % sur des sapeurs-pompiers volontaires, et de conforter leur engagement de volontariat. Ainsi, l'article 23 clarifie la notion d'accident de service pour une meilleure prise en charge des sapeurs-pompiers volontaires par la sécurité sociale. L'article 24 permet aux sapeurs-pompiers volontaires de bénéficier de dons de jours de congé et l'article 22 prévoit un abaissement de cinq ans de la durée d'engagement ouvrant droit à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Je me félicite que le Sénat ait renforcé cette démarche. Nos collègues rapporteurs ont réécrit l'article 30 afin de faciliter l'attribution du label employeur partenaire des sapeurs-pompiers » et d'améliorer le mécanisme de réduction d'impôt au titre du mécénat en lui préférant un dispositif de réduction de cotisations sociales patronales, déjà adopté

Monsieur Pla,

pour les sapeurs-pompiers volontaires justifiant d'une durée exceptionnelle d'engagement égale ou supérieure à trente ans- ils sont nombreux -, ainsi que les modalités de l'harmonisation du régime de l'allocation de vétérance sur celui de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Par cet amendement, nous souhaitons appuyer l'idée qu'il est nécessaire de valoriser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Nous savons que cette préoccupation est largement partagée sur toutes les travées de notre assemblée ; nous vous invitons donc à l'adopter.

Mme Laurence Harribey. L'article 23 tend à confier à l'Association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance la mission de gérer le compte d'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires. Serait ainsi confiée à cette association la collecte des informations nécessaires au traitement des droits à formation ouverts aux sapeurs-pompiers volontaires au titre du compte d'engagement citoyen, ainsi que la collecte des ressources destinées au financement de ces droits,

des informations nécessaires au traitement des droits, d'une part, et de recouvrement des contributions au compte d'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux et intercommunaux de leur ressort, d'autre part. En commission, les rapporteurs ont sollicité le retrait

(APFR) la collecte des informations et des ressources nécessaires à la mise en oeuvre du compte d'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires. Toutefois, une réelle difficulté matérielle se

relatives aux sapeurs-pompiers volontaires qu'ils doivent fournir à l'APFR. Or l'article 23 précise que les communes et les EPCI doivent fournir ces informations lorsqu'ils sont autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires en cause. C'est notamment le cas des corps communaux qui vont être inclus dans les services territoriaux d'incendie et de secours. Dans de tels cas, ce sont bien les communes et les EPCI qui disposent des informations relatives à leurs sapeurs-pompiers volontaires

La réponse des rapporteurs nous satisfait ; nous retirons notre amendement,

nous sommes totalement opposés aux moyens qui sont proposés à cette fin. Et nous sommes navrés qu'il faille en arriver à proposer des dons de congés entre collègues pour défendre les pompiers volontaires Il nous semble que le rôle des congés payés n'est en rien de financer l'engagement et la disponibilité des pompiers. Nous ne pouvons accepter une telle atteinte au droit à congés des salariés : nous pensons qu'il y a là, au fond, une remise en cause camouflée derrière une bonne intention. Adopter un tel dispositif, c'est mettre en avant une solidarité individuelle, une atomisation de ce qu'est réellement la solidarité collective au lieu de recourir à la responsabilité des employeurs et de l'État. Valoriser le volontariat, c'est accorder des droits nouveaux aux pompiers volontaires afin qu'ils puissent s'engager dans leur mission sans se soucier des conséquences sur leurs jours de congé. Nous demandons donc la suppression de cet article : tout simplement, il s'agit là d'une fausse bonne idée.

personnelle, la commission a jugé pertinent de créer un mécanisme similaire pour les sapeurs-pompiers volontaires. Ce don n'est ni culpabilisant, car il est anonyme-

arrive encore trop souvent que les sapeurs-pompiers volontaires aient des difficultés à être libérés par leur employeur, qu'il soit public ou privé. L'objet de cet amendement est donc de faciliter la mobilisation de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant un événement exceptionnel tel que celui que nous avons vécu cet été.

des difficultés. Néanmoins, le code de la sécurité intérieure précise déjà explicitement que seules les « nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou du service public » peuvent justifier le refus de délivrer une autorisation d'absence. Celles-ci sont donc ouvertes sans limitation de durée et concernent les missions de secours et de protection au sens large. En matière de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires le droit existe, il suffit de l'appliquer. La commission demande le retrait de cet amendement.

l'avis de la commission ? Ces amendements visent à instaurer une autorisation d'absence pour les sapeurs-pompiers volontaires de huit jours par année civile et de cinq jours pour les sapeurs-pompiers travaillant dans des PME. ainsi à reprendre le régime en vigueur pour les réservistes opérationnels depuis la loi de programmation militaire pour 2019-2025. Pour autant, il convient de prendre en considération les éventuels effets dissuasifs de cette mesure pour les employeurs en raison des conséquences que ces jours chômés pourraient avoir sur l'activité de leur structure.

Mme Toine Bourrat. Cet amendement vise à favoriser l'accès des sapeurs-pompiers volontaires au logement social en prévoyant des objectifs d'attribution, à l'image du dispositif récemment adopté à l'égard des personnes exerçant une activité professionnelle dans un secteur essentiel.

Les sapeurs-pompiers volontaires, qui assument à la fois des missions de secours et de soin, dont la crise sanitaire a rappelé le caractère indispensable, doivent être inclus dans ce dispositif. Eu égard au caractère indispensable du volontariat, qui concerne 79 % du corps des sapeurs-pompiers français et sur lequel repose l'essentiel de notre modèle de protection civile, il apparaît juste et proportionné de favoriser l'engagement par l'amélioration des conditions matérielles et logistiques de nos volontaires en les intégrant au dispositif susnommé. Quel est l'avis de la

de la Nation. Les sapeurs-pompiers ont évidemment vocation à entrer dans ce cadre. Nous souhaitons que le dispositif prévu dans le projet de loi 3DS puisse être privilégié. Dès lors, il ne nous paraît pas souhaitable de modifier la proposition initiale de cet article, au risque d'avoir deux dispositions

La parole est à Mme Elsa Schalck. L'article 26 vise à exempter de cotisations ordinales certains professionnels de santé retraités et engagés par ailleurs en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Les associations agréées de sécurité civile- la Fédération nationale de protection civile, la Croix-Rouge française, la Fédération française de sauvetage et de secourisme -comptent près de 200 000 bénévoles en France et apportent leurs concours chaque jour aux secours d'urgence, en mettant à disposition leurs compétences et leurs équipements, en formant des milliers de nos concitoyens aux gestes de premiers secours, mais également en assurant la sécurité de centaines d'événements sportifs, culturels et associatifs qui se tiennent sur les territoires de nos communes. Elles remplissent ainsi, aux côtés de l'ensemble de la chaîne du secours, des actions de sauvegarde indispensables, mais aussi et surtout bénévoles. Leur rôle s'est particulièrement vérifié par leur forte mobilisation durant la crise sanitaire de la covid-19. Cet amendement vise dès lors à étendre la disposition prévue à l'article 26 aux bénévoles des associations agréées de sécurité civile afin de les encourager et de les intégrer en tant qu'acteurs à part entière de la sécurité civile, en en reconnaissant l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui partagent un engagement sans faille au service de la Nation, mais aussi des compétences et un dévouement du plus haut niveau. Cette proposition d'ajustement du texte, formulée par la Fédération nationale de protection civile vise à soutenir également ces forces vives dans leurs actions, et à ainsi faire bénéficier de ces dispositions

Tout l'objet de cette proposition de loi vise à mieux reconnaître et récompenser l'engagement des bénévoles de la sécurité civile. Néanmoins, le dispositif d'exonération de cotisation ordinale proposé concerne exclusivement les sapeurs-pompiers volontaires et il n'est pas garanti qu'il puisse s'appliquer tel quel

l'avis du Gouvernement ? Au-delà des arguments de la commission avec lesquels le Gouvernement est en phase, je rappelle qu'une telle disposition instaurerait une rupture d'égalité entre les différents professionnels qui sont inscrits au tableau d'un ordre. Cela nous semble problématique. Avis défavorable.

pas justement de valoriser l'engagement citoyen ? Le volontariat dans la protection, particulièrement quand il s'agit de jeunes lycéens, est un engagement citoyen fort.

des jeunes sapeurs-pompiers s'entend aussi quand il s'agit d'apprécier la validation des acquis de l'expérience, utile dans un parcours de formation continue. Cette précision fait également écho à l'article L. 613-5 du code de l'éducation qui prévoit que « les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur une mesure de bon sens que de faire bénéficier d'un dispositif avantageux ceux qui s'engagent comme sapeurs-pompiers. Quel

Pour autant, le cadre de la validation des acquis de l'expérience ne semble pas convenir à cette fin. Je rappelle que cette procédure offre la possibilité d'obtenir une partie ou la totalité d'un diplôme à condition de justifier au minimum d'une année d'expérience professionnelle

(BNJSP) peut d'ores et déjà bénéficier de la reconnaissance de ce diplôme lors de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire ou de son recrutement en tant que sapeur-pompier professionnel par le biais d'une dispense de formation. Par ailleurs, cette demande sera satisfaite dans le cadre des démarches de certification engagées par la (DGSCGC). J'ajoute que la validation des acquis de l'expérience est soumise à la présentation d'un mémoire et à un passage devant un jury, qui peut également apprécier que des activités non professionnelles,

dans le cadre de leurs activités d'encadrement de jeunes sapeurs-pompiers (JSP). Les sapeurs-pompiers pourront ainsi être considérés en service en cas d'accident ou de maladie contractée à l'occasion de cette activité. Je rappelle le rôle très important des éducateurs qui encadrent les jeunes sapeurs-pompiers. Ils sont bien sûr indispensables pour mettre en place des sections de JSP. l'amendement n° 90. L'article 29 prévoit que l'engagement comme jeune sapeur-pompier et l'obtention du brevet national de jeune sapeur-pompier soient reconnus lors de l'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou dans le cadre du parcours scolaire. On ne peut que souscrire à l'objectif de cette nouvelle mesure. Cet article s'inscrit en cohérence avec l'article 23 de la proposition de loi, qui vise à compléter la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires afin de préciser que ces dispositions sont applicables, quelle que soit la cause de l'accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité de sapeur-pompier volontaire ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal. Il permet également de viser les sapeurs-pompiers professionnels, en cohérence avec la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le présent amendement, par son caractère générique, vise à apporter

employeur partenaire des sapeurs-pompiers » à tout employeur public ou privé ayant conclu une convention de disponibilité avec un SDIS. Ces conventions, prévues à l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, permettent de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Le label acquiert ainsi une valeur législative. Cet article prévoyait également que les entreprises s'étant vu attribuer ce label soient accompagnées par les SDIS pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt figurant à l'article 238 du Plusieurs amendements votés en commission des lois ont supprimé ces dispositions pour les remplacer par un dispositif plus ambitieux : l'exonération de charges patronales, sur le modèle de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. L'exonération va donc s'appliquer pour les sapeurs-pompiers qui sont rémunérés jusqu'à 1,6 SMIC durant cinq ans et avec un double plafond

Il faut également se souvenir que le but fondamental de la commande publique est de permettre à un acheteur public de satisfaire un besoin ou d'exercer une compétence. Chaque fois que l'on s'éloigne de ce principe, c'est le contribuable ou l'usager qui paie la différence. En outre, les dispositions proposées ne semblent pas conformes à l'article 20 de la directive

Les questions de leadership dans la prise de décision ou d'organisation sur le long terme d'une telle plateforme unique doivent s'accompagner d'une réflexion accrue sur les mécanismes de financement et de compensation. d'aide médicale urgente (SAMU) organisent les sorties d'urgence des pompiers pour répondre aux appels, ils deviennent responsables d'une dépense départementale. À l'inverse, si les pompiers sont chargés de faire sortir les véhicules du SAMU dans le cadre de cette expérimentation, ils engagent une dépense ne relevant plus de leur budget. En dehors de ces guerres de clochers, la responsabilité des dépenses devrait aussi être abordée en amont de cette expérimentation. Enfin, ce numéro unique ne doit pas cacher les difficultés de l'aval.

Lors de la discussion générale, nos rapporteurs ont clairement précisé leur souhait de réduire la durée de l'expérimentation de trois ans à deux ans, ce à quoi nous souscrivons totalement.

l'urgence. Aucune évolution ne sera possible tant que l'État ne s'impliquera pas au plus haut niveau et tant que chacun des deux ministères concernés, celui de l'intérieur et celui de la santé, s'obstinera à jouer sa propre partition au nom des différences de culture. Alors que les professionnels de la santé et de la sécurité civile peuvent s'entendre sur le terrain, une volonté de travailler ensemble est absente au niveau national. L'enjeu est pourtant simple : il s'agit de l'optimisation de l'usage des moyens, seule à même de préserver la qualité du service public. Une plus grande efficacité et un meilleur emploi des moyens consacrés au secours passent nécessairement par des coordinations renforcées et des mutualisations élargies. À travers nos échanges sur cet article 31, groupe souhaite obtenir l'assurance que le Gouvernement entend bien procéder à la mise en oeuvre de plateformes départementales, regroupant le 15 et le 18, et non de plateformes supradépartementales, voire régionales, comme le prévoit le projet Marcus.

qui vise à instituer un numéro unique des services d'incendie et de secours. L'expérimentation annoncée ne doit pas masquer les inconséquences manifestes du projet.

D'ailleurs, les assistants de régulation médicale du 15 se sont mis en grève dans une quarantaine de SAMU à la suite de l'annonce de ce projet. Ensuite, les départements, qui assurent la plus grande part du financement des SDIS, souhaitent légitimement avoir la maîtrise des moyens engagés lors des interventions pour en contenir les coûts, ce qui ne serait pas le cas avec la mesure

il me paraît malvenu, sans concertation préalable et dans un contexte juridique et financier plutôt mal ficelé, d'envisager l'expérimentation telle qu'elle est proposée.

en effet à supprimer l'article 31 de la proposition de loi, qui crée un cadre pour expérimenter des plateformes communes de réception des appels d'urgence en vue de la mise en place d'un numéro d'appel unique. Les arguments développés par l'auteur de l'amendement sont audibles, mais nous continuons de penser que des plateformes communes et un numéro unique sont des avancées nécessaires. Néanmoins, nous estimons que les conditions ne sont pas réunies pour les généraliser aujourd'hui. En outre, il ne suffira pas d'un coup de baguette législative pour créer ces plateformes à l'échelle de chaque département. Un important travail de fond et de préparation est nécessaire. C'est la raison pour laquelle l'expérimentation proposée à l'article 31 est, selon nous, un compromis acceptable,

n'est pas une nécessité requise par l'Union européenne, contrairement à ce qui a été dit, mais simplement une recommandation en faveur des expatriés en Europe. Ce n'est pas nécessairement une solution efficace du point de vue de la bonne gestion des moyens de réponse aux urgences, notamment sous l'angle sanitaire. Je ne suivrai toutefois pas la formule de notre collègue, car il existe déjà des situations d'organisation partagée sur un site unique, dans lesquelles les inconvénients

d'urgence déclenche en général une dépense publique qui peut être tout à fait substantielle. Au regard de l'analyse de la qualité des réponses et de l'efficacité de l'orientation des appels,

Cette singularité présente des atouts et des avantages- nous en parlons depuis hier, en particulier pour ce qui concerne le volontariat des sapeurs-pompiers. Mais le modèle de sécurité publique à la française présente aussi des failles et des limites

Cela fait désormais une dizaine d'années que les gouvernements successifs esquivent le sujet, « se défilent » et renvoient la responsabilité à leurs successeurs. Si le traitement de ce sujet est régulièrement renvoyé aux calendes grecques et si l'on multiplie les expérimentations, c'est, me dit-on, pour ménager les susceptibilités des uns et des autres.

de la commission ? Le présent amendement tend à revenir à la version initiale de l'article 31, qui prévoyait la création généralisée de plateformes communes et la mise en place du 112. Pour les motifs évoqués lors de l'examen de l'amendement précédent, et la raison l'emportant, nous sommes contre cette rédaction.

: La parole est à Mme la ministre déléguée. La généralisation des plateformes communes d'appel d'urgence, qui regroupent les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente au niveau national, induit de profonds impacts en termes de gouvernance, de territorialité, de doctrines, de systèmes d'information et de processus métier. Compte tenu de la sensibilité de ce sujet, le Gouvernement estime préférable de rétablir la issue des travaux préalables et des votes de l'Assemblée nationale, en raison des équilibres qui ont été précédemment trouvés sur cet article. L'amendement

L'amendement n° 49 rectifié tend à réintroduire la mention du 112 dans les termes de l'expérimentation. Nous savons que cet ajout n'est pas consensuel, alors qu'il ne change rien à la teneur de l'expérimentation. Nous ne souhaitons pas

de Mme Guidez tend à mentionner que l'expérimentation sera mise en place en lien avec l'association départementale des transports sanitaires urgents. Or le dispositif prévu par l'article fixe déjà comme objectif de faciliter et d'accélérer l'accès aux SAMU. La déclinaison réglementaire de l'expérimentation pourra prévoir une consultation de l'association départementale des transports sanitaires urgents,

de la commission des lois ; l'avis est logiquement défavorable. Cependant, nous ne pouvons que nous interroger, madame la ministre. Comment justifier que l'on écarte les associations agréées de sécurité civile du dispositif, alors que leurs bénévoles jouent un rôle fondamental auprès de nos concitoyens ? Il s'agit là d'une grande injustice à leur Comment mettre en place des expérimentations à l'échelle supradépartementale, alors que le département est l'échelle d'action de la sécurité civile et des SDIS ? Ce serait donc aux acteurs locaux de s'adapter à l'échelle des ARS, alors qu'il serait beaucoup plus simple et efficace de faire l'inverse Comment réintroduire l'expérimentation du regroupement du 15 et de la permanence des soins, alors qu'une telle expérimentation ne concerne en rien la sécurité civile ? Cette mesure est étrangère à ce texte. Elle ne concerne que la santé et devrait avoir sa place dans un texte qui concerne non pas la sécurité civile, mais la santé. Enfin, comment pouvez-vous exclure les présidents des conseils d'administration des SDIS du pilotage de ces expérimentations, alors que celles-ci vont concerner leurs personnels et leurs moyens ?

Si l'expérimentation proposée dans cet article est une étape essentielle et indispensable pour atteindre l'objectif d'un numéro unique d'appel d'urgence, il faut cependant préciser certains aspects relatifs à son application. Tout d'abord, comme l'a dit Olivier Cigolotti, la plateforme doit être absolument départementale. L'amélioration de la prise en charge des personnes étant le point central de l'expérimentation, il est important que la gestion des appels et les décisions prises en matière de santé face à l'urgence de la situation restent entre les mains du médecin régulateur. Il ne peut pas y avoir deux ou plusieurs médecins lors de l'appel en rapport avec la santé, au risque de perdre en efficacité durant l'intervention.

en cause les prérogatives du médecin régulateur. Les plateformes existantes se sont d'ailleurs constituées à droit constant et ne semblent pas avoir remis en cause les fondamentaux de la régulation. Dans l'hypothèse où un modèle de plateforme serait pérennisé, la commission a souhaité préciser que le référentiel de fonctionnement des plateformes devrait notamment garantir le respect du secret médical et qu'il ne remettait pas en cause la mission de régulation médicale ni le service d'accès aux soins.

notamment. Cependant l'Assemblée nationale a fait marche arrière et a remplacé ce dispositif par une expérimentation de plateforme commune de réception des appels d'urgence, avec plusieurs configurations possibles. Des interrogations demeurent quant à cette expérimentation, laquelle se ferait au niveau laquelle se ferait au niveau départemental. Malgré des modifications effectuées en commission des lois, cet article reste finalement assez peu clair sur l'organisation des expérimentations et leur objectif final. Un point nous a particulièrement étonnés, et des collègues élus des départements concernés

d'activité de ces plateformes. D'autre part, nous souhaitons préciser que ces plateformes préexistantes seront associées aux départements nouvellement expérimentateurs. Une expérience de terrain doit être prise en compte, et il semble logique que l'on s'en serve. Tel est le sens de cet amendement, qui exprime également la volonté d'inclusion des acteurs de la sécurité civile déjà engagés sur ces plateaux, notamment dans le projet NexSIS 18-112 qui se développe en parallèle.

des nombreuses plateformes communes de réception des appels d'urgence déjà existantes. Je veux rassurer Mme Brulin : Loïc Hervé et moi-même nous sommes personnellement déplacés à Annecy afin

Cet amendement est contraire à la position de la commission. Il tend à ce qu'un décret précise les modalités et les conditions d'accès aux marchés publics des SDIS, afin de garantir afin de garantir la protection des données de santé et d'autres données personnelles dans le cadre des opérations de secours et d'urgence. Le problème du secret médical est, il est vrai, très sensible. Toutefois, la protection de ces données ne passe pas nécessairement par des adaptions au droit commun de la commande publique, mais plutôt par les normes et agréments qui s'appliquent aux dispositifs et instruments médicaux pour autoriser leur utilisation

pour des raisons que chacun comprendra, à toutes les actions entreprises par les services d'incendie et de secours de l'État. Je puis vous assurer que la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en lien étroit avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), accompagne les SDIS dans le renforcement de leurs dans le renforcement de leurs pratiques et des outils en matière de sécurité des systèmes d'information. Le futur système de gestion de l'alerte NexSIS, qui est développé par l'Agence du numérique de la sécurité civile et qui a vocation à être déployé dans l'ensemble des SDIS, bénéficie également de cette sécurité des systèmes d'information conçue nativement grâce à l'expertise des cadres du ministère de l'intérieur, que je veux saluer. La détermination par décret de l'accès des modalités et des conditions d'accès aux marchés publics des SDIS, afin de garantir la protection des données de santé et des autres données personnelles dans le cadre des opérations de secours et d'urgence, ne nous apparaît donc pas nécessaire. Je vous propose donc de retirer cet amendement.

précisant les conditions dans lesquelles seront accueillies et traitées les données transitant par ce numéro unique. Actuellement, des situations justifient clairement

Cet amendement est contraire à la position de la commission. Il est relativement proche de l'amendement précédent, à la réserve près qu'il ne s'inscrit pas au sein des dispositions expérimentales. J'en demande le retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.

SDIS. La Cour des comptes l'a relevé : comment expliquer que cette agence pratique un taux d'internalisation de seulement 5,8 % au lieu des 37 % recommandés, et externalise donc plus de 94 % de ses activités, de grandes entreprises extraeuropéennes comme l'américaine Google ou la qatarie Inetum ? La question de la souveraineté numérique ne peut être ignorée face aux risques d'utilisation dérivée d'un certain nombre de données personnelles. Comme les collectivités financent 83 % de ce projet vers lequel la dotation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours de 2020 a été entièrement ces interrogations sont légitimes et nous attendons des réponses. La proposition de loi contient déjà plusieurs demandes de rapport, en particulier à propos de la réforme de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et des aides aux employeurs pour le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires.

et de la sécurité civile NexSIS 18-112 pour un vice de forme tenant au défaut de consultation de l'autorité de la concurrence a conduit à la publication d'un nouveau décret le 21 juillet 2021, sans menacer ou impacter le développement de l'outil. L'avis du

L'article précise bien que la création d'une réserve constitue une faculté et non une obligation, mais nous jugeons utile de préciser dans la loi que la création des réserves ne puisse pas se faire au détriment des Unions départementales associatives.

comprenons la volonté de ne pas créer une réserve citoyenne au détriment des associations agréées de sécurité civile existantes. Néanmoins, nous ne pensons pas que le mécanisme proposé soit efficace,

à Mme la ministre déléguée. Cet amendement vise à étendre la possibilité de création de réserves citoyennes des services d'incendie et de secours à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.

dont de nombreux infirmiers. L'article 33 de cette présente proposition de loi instaure la possibilité pour les étudiants en santé d'effectuer un stage au sein d'un service départemental, et je tiens à saluer cette disposition. Dans le département de la Haute-Garonne, nous expérimentons depuis déjà plusieurs années la possibilité pour les étudiants en médecine, pharmacie ou en soins infirmiers de faire des stages au sein du SDIS. À la suite d'un récent accord avec le doyen de la faculté de médecine de Toulouse, les

Ces stages peuvent aussi être l'occasion d'un terrain de recherche en médecine d'urgence et en médecine du travail pour les étudiants en thèse. Ils peuvent ainsi faire évoluer la pratique médicale d'urgence dans notre pays.

sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. En pratique, les infirmiers représentent la majorité des effectifs au sein des services de santé et de secours des SDIS- sachez que, en 2019, ils étaient deux fois plus nombreux que les médecins, et quatorze fois plus nombreux que les pharmaciens. Cet amendement du groupe RDPI s'inscrit donc dans les recommandations des rapporteurs de la commission des lois, et tire toutes les conséquences de cet état de fait, en proposant d'étendre ces stages aux étudiants des instituts de formation de soins infirmiers.

Ce dispositif ne semble pas nécessairement relever du niveau législatif, et son inscription dans le code de la sécurité intérieure ne me semble pas adéquate. Le présent amendement tend, d'autre part, à préciser que le règlement opérationnel pris par le maire ou le préfet pour l'emploi des moyens des SDIS prévoit aussi les conditions d'emploi des associations agréées de sécurité civile. Cette précision semble inutile, puisque l'article 725-3 du code de la sécurité intérieure tel que propose de le modifier l'article 34 notre amendement prévoit déjà les conditions d'emploi des associations agréées

Cet amendement vise à conforter le rôle et les missions des associations agréées de sécurité civile, dans lesquelles elles s'engagent pleinement avec leurs bénévoles et leurs salariés. Compte tenu de ce rôle, la reconnaissance par la Nation de l'engagement des bénévoles de ces associations agréées est également clairement rappelée. Enfin, nous rappelons par cet amendement que les associations agréées sont également engagées par conventions, en cohérence avec les modifications portées à l'article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure.

à M. Christian Redon-Sarrazy. Nous proposons de clarifier les conditions d'emploi des associations agréées dans le cadre des opérations de mise en oeuvre du plan Orsec, en les intégrant à la chaîne de commandement constituée par le directeur et le commandant des opérations de secours. des opérations de secours. Dans le cadre des opérations du plan Orsec, les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la participation des associations agréées s'inscrivent dans le règlement du code général des collectivités territoriales, et ces associations sont effectivement placées sous l'autorité du directeur et du commandant des opérations de secours.

l'avis de la commission ? Les modalités de participation des associations agréées de sécurité civile ont davantage vocation à être détaillées dans le plan Orsec lui-même que dans le règlement opérationnel arrêté par le préfet. Le code de la sécurité intérieure prévoit d'ailleurs déjà la fixation au sein même des plans Orsec départementaux et zonaux des conditions d'emplois des moyens par les autorités compétentes pour diriger les opérations de secours.

Si l'on peut se féliciter de l'élargissement par le présent article des cas dans lesquels une personne morale de droit public pourra se constituer partie civile en cas d'incendie volontaire, il nous paraît nécessaire, par esprit de cohérence, d'étendre cette possibilité aux incendies involontaires, car les moyens matériels et humains engagés sont identiques. est l'avis de la commission ? Faire peser la charge financière de l'extinction d'un incendie sur l'auteur d'un incendie involontaire sans qu'il s'agisse formellement d'une sanction pénale conduirait à lui faire subir une pénalité financière que nous jugeons excessive par rapport à la gravité de l'action qu'il a pourtant

dont la responsabilité échoit aux maires, peuvent participer au financement de l'allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal.

La rédaction proposée par l'Assemblée nationale englobe d'ores et déjà les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les marins-pompiers. Les auteurs de cet amendement proposent d'inclure dans cette disposition nécessaire et protectrice les agents relevant des filières administratives et techniques

Cet ajout nous semble inutile, puisque le code pénal expose très clairement que l'obligation de porter assistance à un tiers en péril est conditionnée par l'absence de risque pour soi ou pour les tiers. L'ajout de règles voisines dans un autre code risque de nuire à l'intelligibilité de la loi pénale, raison pour laquelle

le texte de la commission, modifié, l'ensemble de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers